Il y avait déjà beaucoup trop de dérogations, mais, avec cette mesure, les 800 000 personnes en situation de handicap, sans compter les enfants ni les personnes vieillissantes en perte d'autonomie, ne pourront plus accéder qu'à quelques milliers de logements neufs chaque année. texte remet en cause le principe de l'accessibilité universelle : « une grave régression sociale », « un recul gigantesque », selon les associations. En réalité, vous cédez au lobby des promoteurs immobiliers, qui réclamaient cette mesure, en faisant d'ailleurs porter indignement le chapeau de la réduction des pièces à vivre à l'accessibilité une contre-vérité au regard d'une tendance beaucoup plus lourde à la réduction de la superficie globale des logements, de l'ordre de 10 % à 15 % en quinze ans. Votre dispositif fait primer le marché sur la solidarité,

se réaliser. Au fond, le logement doit répondre aux besoins de chacun et l'accompagner tout au long de sa vie. Cela n'empêchera nullement une personne à mobilité réduite de rendre visite à quelqu'un dans son appartement, car toutes les parties communes vont rester accessibles, de même que le séjour et les toilettes des logements.

à vivre sous le seuil de pauvreté. En réalité, monsieur le secrétaire d'État, vous créez des citoyens de seconde zone, à rebours des promesses électorales de M. Macron.

la politique de cohésion. Dans un jeu de rôles absolument parfait, le Gouvernement s'y est opposé. Pourtant, voilà quelques jours, le commissaire Oettinger, auditionné au Sénat, soulignait un double jeu de la France. Après avoir laissé entendre, au Conseil européen de février 2018, que la France pouvait être favorable à un redéploiement des fonds européens vers les nouvelles priorités, aujourd'hui on crie au loup et, en même temps- je dis bien « en même temps » -, on bloque les contributions nationales. Comment justifier cette évolution contradictoire ? Comment allez-vous réussir à mener de front la défense de politiques dites de solidarité- PAC, cohésion -, la mise en oeuvre de nouvelles politiques-

vous l'avez dit, la proposition de budget présentée par la Commission n'est qu'un projet. Elle prend en compte les nouvelles priorités qui

auraient une incidence directe sur la viabilité de nombreuses exploitations agricoles. Pour nous, il ne fait aucun doute que la politique agricole commune est au coeur des enjeux stratégiques de l'Union européenne : c'est un élément de notre souveraineté, de notre sécurité alimentaire, ainsi que de notre compétitivité. La PAC permet d'aider l'agriculture à relever le défi de l'environnement et du changement climatique.

pour répondre aux nouveaux enjeux, définir un nouveau modèle agricole et alimentaire et résorber les fractures territoriales. Cela suppose un renouvellement en profondeur et partagé, qui ne peut se résumer à des effets de com'ou à une tarentelle qui va et qui vient. À propos de tarentelle, avant l'improbable coalition populiste en Italie, il y a eu un gouvernement Renzi qui avait beaucoup de points communs avec le nôtre. Prenons garde collectivement de ne pas donner prise à cette évolution en France, à un an des élections européennes. Cela suppose une relation adulte les acteurs de la vie démocratique et une position française clairement énoncée. La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour le groupe Les Indépendants-République et Territoires.

Ce héros est un enfant de La Réunion, même s'il a grandi en Indochine dans une famille d'avocats avant de découvrir la métropole et de se consacrer à la grande passion de sa vie, la mécanique. Fondateur d'une entreprise de voitures, ce jeune homme brillant a surtout été l'un des pionniers de l'aviation française. connaissez tous dans cet hémicycle : Roland Garros. Premier aviateur à traverser la Méditerranée et à relier deux continents, en septembre 1913, Roland Garros n'est pas seulement un aventurier. C'est aussi un inventeur de génie. C'est lui qui, en janvier 1915, a révolutionné l'aviation militaire, avec Raymond Saulnier, en inventant un dispositif de mitrailleuse aérienne. C'est le travail de ces deux hommes qui a assuré à la France la maîtrise du ciel pendant la Première Guerre mondiale. Les noms célèbres de Fonck ou de Guynemer font écho à son engagement au service de la France. Patriote, Roland Garros l'est indéniablement par son engagement héroïque lors des combats aériens de la guerre de 14-18. Monsieur le ministre, il y a un siècle, Roland Garros s'évade d'un camp de prisonniers, de manière rocambolesque, et finit sa course, abattu, le 5 octobre 1918, la veille de ses trente La France a célébré son parcours en lui décernant une citation à l'ordre de l'armée et en donnant son nom à un stade construit dans les années vingt, porte d'Auteuil, où s'affrontent aujourd'hui les plus grands champions internationaux de tennis. Je crois, monsieur le ministre, que Roland Garros mérite aujourd'hui d'entrer au Panthéon.

La France lui doit beaucoup, et la population réunionnaise aimerait vous voir soutenir la proposition que le conseil régional de La Réunion défend depuis avril 2016 et dont l'adoption pourrait symboliser le centenaire de la fin de la Grande Guerre, que nous célébrons cette année.

Dans le domaine de l'éducation nationale, le département bénéficiera à la rentrée prochaine de 466 postes supplémentaires pour le seul premier degré et du dédoublement des classes. Ma collègue garde des sceaux est également pleinement mobilisée pour améliorer la situation au tribunal de grande instance de Bobigny elle s'est engagée à pourvoir l'ensemble des postes de magistrat et de fonctionnaire dès septembre 2018 et à affecter un certain nombre de magistrats en surnombre.

alors qu'elles avaient diminué entre 2010 et 2014, elles sont aujourd'hui au plus haut, et nous avons choisi un premier quartier de conquête républicaine. Nous avons Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler entre nous : peut-être faut-il, concernant la région d'Île-de-France, en particulier la première couronne, engager un certain nombre de réformes de structure. Monsieur le ministre, assez de rapports, assez de visites ministérielles ; des actes ! Le 22 mai dernier, beaucoup d'élus

comment voulez-vous que la politique de la ville donne des résultats, monsieur le ministre ? Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, nous ne sommes pas là pour être visités ! Nous voulons des actes, nous y avons droit, comme partout en France

BNP Paribas ayant explosé tous les scores en payant 8 milliards d'euros à ce titre en 2014, une somme sans précédent. Pour faire simple, utiliser le dollar dans les transactions ou même avoir une adresse e-mail dont le serveur est situé aux États-Unis suffit pour être poursuivi. La France n'est pas le seul pays européen dans cette situation, bien entendu, les Allemands étant logés à la même enseigne. Aujourd'hui, le chantage pèse sur nos entreprises actives en Iran. PSA, Total et d'autres s'apprêtent à quitter le pays, alors que les Japonais et les Chinois y restent.

historiques obtenus grâce à cet accord en matière de non-prolifération nucléaire. Cela étant, nous sommes conscients des incidences économiques importantes que peut avoir le retour des sanctions américaines pour les intérêts des entreprises françaises et européennes, et européennes, les décisions restant prises par les opérateurs économiques et les entreprises. Pour les accompagner, notre stratégie s'appuiera sur une double approche. À court terme,

à cette situation asymétrique. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et Bruno Le Maire sont convenus de travailler sur des dispositifs permettant de renforcer l'indépendance économique de l'Europe. Nous avons ainsi engagé des travaux, en France et avec nos partenaires européens, pour développer des outils permettant de mieux protéger nos entreprises contre l'extraterritorialité des sanctions américaines. C'est l'objet de la révision du règlement européen de 1996 dit « de blocage », qui vise à offrir un dispositif plus protecteur pour nos entreprises et plus dissuasif à l'égard des autorités étrangères. La Commission européenne a proposé hier des amendements nécessaires. Nous soutenons cette approche.

Le troisième axe d'action serait de donner à l'Union européenne la capacité de dialoguer d'égal à égal avec les États-Unis, et donc de réfléchir à un équivalent européen de l'américain. Il y a encore

Pour dynamiser ces lycées, il a annoncé des mesures d'importance, dont deux qui rapprochent les lycées du monde de l'alternance. La première est la création de campus d'excellence. Ces campus, au nombre de trois par région, et le dynamisme qu'ils dégageront sauront susciter l'envie et motiveront les jeunes. et motiveront les jeunes. Ils comprendront des établissements proposant des filières professionnelles allant du CAP à la licence, un internat, des infrastructures sportives et culturelles, des incubateurs d'entreprises, mais aussi des centres de formation d'apprentis. La seconde mesure est la création, dans chaque lycée professionnel, d'unités de formation en apprentissage. Les jeunes pourront ainsi confronter leurs expériences, passer d'une filière à l'autre sans remettre en cause leur cursus, appréhender d'une manière plus sereine le monde de l'entreprise. L'objectif est clair : créer des synergies entre les formations initiales et l'alternance. Pour autant, ne faudrait-il pas aller plus loin ? Ne serait-il pas pertinent plus loin ? Ne serait-il pas pertinent de lisser les heures de cours sur les trente-six semaines d'enseignement pour les professeurs de formations initiales ?

Différents leviers sont mobilisés pour cela, mais il est essentiel que nous puissions promouvoir l'innovation pédagogique et la personnalisation des parcours ; c'est le sens de la proposition que vous avez formulée. Il faut

de la santé ... La France compte 1,5 million de personnes de 85 ans et plus. À l'horizon de 2050, elles seront près de 5 millions. La question de la dépendance est donc aujourd'hui cruciale.

Le profil des populations accueillies en établissement a évolué : les résidants souffrent de pathologies multiples, de maladies chroniques et dégénératives. Dans ce contexte, les professionnels doivent faire face à des conditions de travail difficiles : le manque d'effectifs et de temps est régulièrement et légitimement mis en avant. a annoncé la semaine dernière des mesures en faveur des EHPAD, avec pour objectif l'amélioration « dans l'immédiat de la qualité de vie des personnes âgées » et l'anticipation de la perte d'autonomie. Cette feuille de route a permis de rassurer, mais ne règle pas tous les problèmes. En effet, de nombreux EHPAD rencontrent des difficultés en matière de recrutement, qu'il s'agisse des aides-soignants, des infirmiers, des médecins coordinateurs ou des directeurs. Le personnel en place est donc confronté à des cadences infernales, à un et à un absentéisme importants et à un taux d'accidents du travail deux fois plus élevé que la moyenne nationale. On ne peut que constater le manque d'attractivité du secteur des personnes âgées, réputé difficile, mal payé et mal considéré, faute de ressources suffisantes pour améliorer les conditions de travail dans des métiers pénibles physiquement et psychologiquement. Des directeurs assument souvent la responsabilité de plusieurs établissements, par intérim, pendant de nombreux mois, voire des années. À titre d'exemple, dans le département du Puy-de-Dôme, sur les vingt-six établissements publics autonomes, plus d'une dizaine ont une direction temporaire. Ces modes de gouvernance sont préjudiciables au bon fonctionnement et à la modernisation des structures. Pourtant, notre société doit relever ce défi de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. Quelles sont les mesures prévues par le Gouvernement pour favoriser le recrutement pérenne de directeurs et, plus largement, pour rendre les métiers liés à la dépendance plus attractifs ? La parole

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a pris et continuera de prendre ses responsabilités. Premièrement, nous débloquons d'importants moyens financiers : les EHPAD recevront 360 millions d'euros supplémentaires de 2019 à 2020 pour recruter des personnels soignants. La généralisation

un changement de tarification, pourtant inspiré par une bonne intention, a eu comme conséquence d'affaiblir financièrement près d'un tiers des EHPAD ; il convient de neutraliser cela. Troisièmement, nous entendons agir sur les conditions de travail du personnel, en améliorant le matériel, les techniques de management et l'accompagnement du personnel. Dans les années à venir, nous devrons définir,

a présenté ce qu'elle a appelé les grandes orientations de la réforme de l'audiovisuel public. Malheureusement, les annonces faites ne sont à la hauteur ni des enjeux ni des attentes de l'ensemble du secteur. Si certaines annonces vont dans le bon sens- je pense notamment à la sanctuarisation financière de la création, qui sera, je l'espère, effective, à l'investissement dans le numérique, qui doit permettre de répondre aux attentes du jeune public, ou encore au recentrage de la mission de France 3 sur la proximité -, la volonté manifeste du Gouvernement de réaliser des coupes budgétaires alors que le service public audiovisuel français est déjà sous doté ne démontre pas une grande ambition pour celui-ci ...

Outre ces suppressions, il est à craindre que les réductions budgétaires envisagées, ainsi que la transformation de l'organisation des sociétés, n'entraînent des plans de licenciement. Le financement et la gouvernance sont les grands absents de la présentation. Monsieur Castaner- j'imagine que c'est vous qui allez répondre à ma question -, pourriez-vous nous indiquer comment le Gouvernement compte atteindre ses objectifs ? Par ailleurs, quelles sont les ambitions du Gouvernement pour l'audiovisuel extérieur, qui devrait faire l'objet d'une réflexion ?

Cette décision a choqué celles et ceux qui attachent de l'importance aux questions environnementales, notamment à la déforestation. D'ailleurs, la réponse agacée de M. Hulot la semaine dernière devant notre assemblée est révélatrice d'une véritable incohérence. Si je m'adresse au ministre de l'agriculture, c'est que, au-delà du renoncement écologique, apparaît une réelle absence de cap pour l'agriculture française. Alors que les filières colza et tournesol sont en mesure de produire la matière première des biocarburants, vous avez délibérément privilégié l'huile de palme. Alors que M. Hulot nous a imposé, il y a quelques mois, l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures sur le sol français,

ont aujourd'hui besoin non seulement de l'attention de l'État, mais aussi d'une véritable stratégie agricole française

Ce projet a été décidé en 2015, à la demande du gouvernement précédent, pour mettre en place une solution de reconversion d'un site pétrolier et sauver ainsi 250 emplois. Les syndicats agricoles invitent à une mobilisation à compter de dimanche et envisagent le blocage de treize raffineries. Je comprends la préoccupation qui est la vôtre et qui est également celle des agriculteurs. J'en appelle néanmoins à l'esprit de responsabilité pour éviter de pénaliser nos concitoyens et nos entreprises, qui seraient les premiers touchés par un blocage des raffineries. Ce blocage toucherait le monde agricole lui-même, qui souffre déjà des difficultés actuelles du transport ferroviaire. L'approvisionnement de l'usine de La Mède pourra évoluer au fil du temps pour intégrer davantage de matières agricoles françaises : c'est possible et souhaitable, car les contrats qui pourraient être conclus dans la durée avec les filières françaises seraient créateurs de valeur et sources d'emplois sur le territoire national. La parole

Union Centriste. Ma question s'adressait à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Samedi dernier, une marche blanche s'est déroulée à Bourges, sur l'initiative du corps médical et en présence de nombreux élus, dont le président de la région Centre-Val de Loire.

À l'hôpital de Blois, les services se dégradent et des réaménagements sont nécessaires par manque de personnel et d'entretien ; il n'y a qu'une douche pour tout un service Cela fait plusieurs mois que cette crise dure. En avril, le conseil régional a refusé à l'unanimité de valider le projet régional de santé présenté par l'ARS.

Le manque de personnel soignant dans la région et la désertification médicale représentent un problème majeur, qui perturbe gravement le fonctionnement des services de santé, quand il n'entraîne pas leur fermeture pure et simple, comme pour la maternité de Châteaudun. Désormais, les parturientes doivent se rendre dans les autres maternités de la région, la plus proche étant à Alors que M. le Président de la République s'apprête à présenter une réorganisation du système de soins, un rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie publié mardi préconise la création d'établissements de santé communautaires de proximité.

Des efforts importants sont demandés à l'hôpital public pour maintenir une offre accessible et de qualité. Il faut que les raisons en soient bien comprises. Je veux d'abord rappeler que la bonne gestion des établissements n'est pas un problème en soi ; elle est même éthique

C'est l'enjeu de la réforme que mène actuellement la ministre des solidarités et de la santé. Elle a renforcé la mission relative à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Le Gouvernement réfléchit également à l'évolution des modèles de financement afin de valoriser davantage la prévention, la qualité et la pertinence

Fin mai, en tant que président du groupe d'amitié sénatorial France-Yémen, j'ai fait partie d'une délégation de parlementaires qui, à l'invitation de la coalition, a pu rejoindre Mareb, enclave « sécurisée » située à deux heures de vol de Riyad. Nous étions accompagnés de l'ambassadeur de France au Yémen. Il faut souligner qu'il s'agit de la première délégation parlementaire à s'être rendue sur place depuis le début du conflit. Je ne m'étendrai pas sur la mauvaise polémique à laquelle a pu donner lieu l'organisation de ce voyage. J'ai pleinement conscience que le contexte de ce pays en guerre et de ce coin du monde appelle à la plus grande prudence. L'Arabie Saoudite compte y jouer un rôle prédominant, sur les plans tant politique que militaire et humanitaire. Nous avons pu nous rendre dans des centres humanitaires, des hôpitaux et des camps de réfugiés. Nous avons notamment visité le centre d'accueil du King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, organisation humanitaire du Gouvernement saoudien dont nous avons rencontré le directeur à Riyad. Ce centre a notamment pour mission d'extraire les enfants soldats de leur condition.

à la grave question du choléra, elles sont extrêmement floues. Dans ces conditions de trouble extrême, quels sont, madame la ministre, vos attentes et vos objectifs en ce qui concerne la conférence humanitaire proposée par le Président de la République pour

la guerre au Yémen dure depuis trois ans. Le conflit est dans l'impasse et le pays est confronté à une triple crise : humanitaire, sanitaire et alimentaire.

Ces obligations s'imposent à toutes les parties au conflit : les rebelles houthis, qui en sont à l'origine, et la coalition arabe, qui est venue au Yémen à l'appel du gouvernement légitime du pays et qui combat aussi Daech et Al-Qaïda. Ces obligations doivent être observées par tous et nous voulons les faire respecter. C'est ce qui a conduit le Président de la République à décider l'organisation d'une conférence internationale humanitaire avec l'Arabie Saoudite. Elle aura lieu à Paris le 27 juin prochain. Il ne s'agit pas d'une conférence de donateurs, les pays de la coalition arabe ayant déjà annoncé 1,5 milliard de dollars d'aide humanitaire pour le Yémen en 2018. Il ne s'agit pas non plus d'une conférence politique, une telle responsabilité revenant aux Nations unies et à leur représentant spécial, dont nous soutenons pleinement l'action.

qui soutient la rébellion et déstabilise cette région.

Je souhaite me faire ici le porte-parole des nombreux élus de Haute-Savoie, mais également d'autres départements, qui subissent des installations illicites de gens du voyage sur le territoire de leur commune et ne disposent que de très peu de moyens pour les empêcher.

Avec mes collègues Loïc Hervé et Jean-Claude Carle et le président de l'association des maires de Haute-Savoie, nous avons maintes fois interpellé les ministres de l'intérieur successifs. Nous avons élaboré une proposition de loi, qui a été adoptée par notre assemblée fin octobre 2017, mais dont le texte a été modifié par l'Assemblée nationale, sans même que son examen le doublement des peines encourues et la possibilité de saisie des véhicules que nous proposions d'instaurer ont été supprimés. Seule la création d'une amende forfaitaire délictuelle très importante a été maintenue.

Madame la ministre, vous devez doter les forces de l'ordre de moyens humains et matériels importants, permettant de faire appliquer les lois de la République durant les périodes d'occupation. Comment expliquez-vous qu'un groupe ayant reçu du préfet une mise en demeure de quitter les lieux soit toujours sur place une semaine après ?

illicite et d'augmenter le quantum de peine. Par ailleurs, une commune respectant ses obligations en matière d'aires d'accueil bénéficiera de la procédure d'évacuation administrative en cas d'occupation illicite, même si son EPCI ne satisfait pas, lui, à ces obligations. C'était là une demande forte des élus. Il faut conclure ! Le Gouvernement continuera à soutenir cette position. Je travaillerai sur ce dossier le 21 juin à l'Assemblée nationale. Il appartient maintenant à chacun de poursuivre cette oeuvre collective.

La séance est reprise. Mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancienne collègue Monique Papon, qui fut sénateur de la Loire-Atlantique de 2001 à 2011. sénatoriale aux entreprises, de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise, présentée par MM. Claude Nougein, Michel Vaspart et plusieurs de leurs collègues

J'en ai malheureusement été trop souvent le témoin dans mon département, la Corrèze. Une entreprise que l'on n'arrive pas à transmettre, c'est un vivier d'emplois qui disparaît, et cela peut porter un coup fatal à un territoire, surtout en zone rurale. En France, nous constatons que la transmission familiale ne concerne que 14 % des cessions de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, ou ETI. C'est l'un des plus faibles taux d'Europe Cette situation suscite des interrogations. Le plus préoccupant, c'est qu'elle se traduit fréquemment par un rachat prématuré par un grand groupe, souvent étranger d'ailleurs. Elle quitte alors très souvent le territoire au bout d'une dizaine d'années. La fermeture de l'entreprise n'est pas la seule conséquence : le déplacement d'un siège social a des répercussions sur tous les services périphériques, qu'ils soient administratifs ou assurés par des professions libérales.

Selon une étude de 2013 de la Direction générale du Trésor, entre 700 000 et 900 000 entreprises ont été ou seront concernées par la reprise entre 2000 et 2020. Ce phénomène va croissant, du fait de l'accélération du vieillissement des dirigeants d'entreprises. En effet, 20 % des patrons de PME sont âgés de plus de soixante ans, et plus de 60 % des dirigeants d'ETI ont plus de cinquante-cinq ans. Nous devons nous préoccuper de l'avenir de ces entreprises qui font vivre nos territoires.

Après avoir auditionné quatre-vingts personnes, nous avons présenté à la délégation un rapport d'information, qu'elle a adopté en février 2017. Il concluait que la modernisation de la transmission d'entreprise était une urgence pour l'emploi dans nos territoires.

transmission, non plus, évidemment, que l'ensemble des autres freins qui persistent à rendre complexes, risquées et coûteuses la transmission et la reprise d'entreprises. La proposition de loi issue de ce rapport a été cosignée par un grand nombre de sénateurs, que je remercie de leur soutien. sous-tendu par l'ambition de répondre aux diverses difficultés que nous avons identifiées. En premier lieu, faciliter la transmission demande de savoir de quoi l'on parle. D'une part, au niveau global, le suivi statistique des cessions et cessations d'entreprises fait défaut. L'INSEE ne serait aujourd'hui pas en mesure d'effectuer ce suivi, ce qui est problématique. Il est essentiel de faire en sorte que puissent être consolidées les données éparses et aujourd'hui non exploitables émanant des tribunaux de commerce, ainsi que de la Direction générale des finances publiques. Il faut également reconnaître à l'INSEE la possibilité d'exploiter les données déclaratives relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés. Sur ces points, madame la secrétaire d'État, j'aimerais obtenir des garanties, car une meilleure connaissance statistique des cessions et transmissions d'entreprises est indispensable pour ajuster la politique publique sur ce sujet. D'autre part, pour chaque opération de transmission, l'information du cédant et du repreneur doit être améliorée. raison pour laquelle le dirigeant doit pouvoir, en toute sécurité, déduire de l'impôt sur le revenu les frais de diagnostic de la transmission de son entreprise. La commission des finances estime que c'est déjà le cas, dès lors que ces dépenses sont effectuées dans l'intérêt de l'entreprise. J'espère que cette interprétation sera bien celle qui sera retenue par l'administration fiscale. Nous souhaitons également encourager les entrepreneurs à anticiper la transmission de leur entreprise et, pour cela, nous proposons d'accroître l'abattement fiscal en cas de donation de parts d'entreprise. En outre, afin d'encourager les jeunes et les actifs à se tourner vers la reprise d'entreprise, nous plaidons pour que la création mais aussi la reprise d'entreprise soient valorisées dans les formations initiale et continue.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, outre les points déjà évoqués par M. Claude Nougein, le texte que nous vous soumettons tend à lever le frein principal à la transmission d'entreprise, à savoir la complexité de son encadrement juridique et fiscal. La France cumule des dispositifs qui, ensemble, peuvent sans doute permettre une transmission à des prix raisonnables, surtout depuis la disparition de l'ISF, mais, pour y parvenir, les entrepreneurs Nous proposons donc de moderniser le « pacte Dutreil », qui prévoit des avantages fiscaux contre des engagements en termes de durée de détention des titres. Notre texte rend plus avantageux le dispositif Dutreil en portant à 90 % le taux d'exonération fiscale, contre un allongement à huit ans de la durée totale des deux engagements. Il assouplit l'obligation de maintien des participations pendant la durée de l'engagement, notamment en cas d'interposition de société entre le redevable et la société éligible au Pour plus de simplicité, nous proposions de supprimer les obligations déclaratives que doivent spontanément observer les donataires, chaque année, pour attester du respect du pacte, sans quoi ce dernier devient caduc. La commission des finances préfère reprendre la rédaction adoptée par le Sénat pour le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance : les obligations déclaratives annuelles seraient maintenues, mais les déclarations devraient être produites sur demande de l'administration. Notre texte permet, en outre, que la donation de titres placés sous engagement individuel puisse se faire à des donataires autres que les seuls descendants, ce qui peut faciliter la transmission à des salariés. Il précise aussi les possibilités d'apport de titres à une et prévoit de mieux définir la notion de animatrice, dont le flou actuel entretient une insécurité juridique qui est la principale source du contentieux dans l'application des pactes Dutreil. Cette proposition de loi tend à améliorer le régime de l'apport-cession, qui n'a que très peu d'intérêt et beaucoup d'effets pervers dans sa version en vigueur : il s'agit de favoriser le réinvestissement dans une PME des produits de cession d'une société. Nous avions également envisagé de proposer une expérimentation pour faciliter la transmission dans deux secteurs auxquels nous sommes très attentifs, l'agriculture et l'artisanat. Il apparaît, à l'examen, que le dispositif soulève des questions, et ce au sein même des professions concernées. Son adoption aujourd'hui nous semblerait donc prématurée, mais nous devrons veiller à revenir sur ce sujet important lors d'un de l'examen texte traitant d'agriculture ou de fiscalité. C'est une attente de la profession agricole, notamment des jeunes agriculteurs. Le dernier chapitre de la proposition de loi répond à l'ambition de favoriser les reprises internes, c'est-à-dire les reprises par les salariés. C'est en effet une possibilité importante de transmission des entreprises qui doit être encouragée. La loi Hamon de 2014, en établissant une obligation rigide d'information préalable des salariés, a fragilisé ce mode de transmission. Le délai imposé est trop court pour permettre aux salariés de s'organiser, tout en étant trop long pour ne pas fragiliser l'entreprise. En effet, les transmissions internes réussies se préparent très en amont et en toute confidentialité. Dans les faits, les dirigeants préfèrent souvent payer la pénalité prévue, plutôt que de respecter l'obligation d'information préalable. C'est un comble vous est soumis vise donc à abroger ces dispositions de la loi Hamon. Les salariés devront cependant toujours être informés de la possibilité de présenter une offre de reprise, mais à un stade où cette information ne risque pas d'hypothéquer les chances d'une reprise en train de se dessiner. Les abattements fiscaux prévus lors d'une reprise par un ou plusieurs salariés seraient relevés de 300 000 à 500 000 euros, et le nombre minimal de salariés-repreneurs requis pour ouvrir droit à un crédit d'impôt en faveur de la société reprise en interne serait réduit de quinze à cinq pour toutes les entreprises comptant plus de quinze salariés.

vingt-sept préconisations ont été très appréciées des entreprises et des professionnels de la cession-transmission. Il a suscité beaucoup d'articles de presse et une proposition de loi qui constitue l'aboutissement de ce travail. C'est une approche globale de la transmission d'entreprise, depuis la TPE jusqu'à l'ETI. Cette proposition de loi permettra d'aider à maintenir les entreprises sur leur territoire et de fluidifier et faciliter les cessions et transmissions, qui sont toujours des moments particulièrement délicats pour nos entreprises. Je ne doute pas que le Sénat soutiendra ce soir

Ce rapport d'information de Claude Nougein et de Michel Vaspart, dont je souhaite souligner ici la très forte implication dans ce travail d'ampleur, met en lumière l'urgence de simplifier la transmission d'entreprise pour maintenir l'emploi sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones rurales.

Les transmissions d'entreprise sont donc appelées à se multiplier en raison des évolutions démographiques. Les difficultés liées à la transmission des entreprises sont identifiées depuis longtemps et ont donné naissance à de nombreux dispositifs fiscaux incitatifs, dont certains peuvent se cumuler.

La proposition de loi dont nous débattons va bien au-delà d'un assouplissement du dispositif Dutreil, puisque les sujets abordés ne sont pas uniquement de nature fiscale. Quatre articles lèvent des freins liés à des complexités du droit du travail ou encouragent la formation vers l'entrepreneuriat. Ces sujets seront abordés par ma collègue Pascale Gruny.

favoriser la transmission des entreprises afin d'éviter leur disparition par rachat, par absorption ou par fusion avec un groupe de taille plus importante et de se donner ainsi toutes les chances de préserver l'emploi et, notamment, son ancrage territorial. Concernant le coût de ce texte pour les finances publiques, nos travaux se sont rapidement heurtés aux lacunes du système d'information statistique. Dans un rapport de mai 2016, l'Observatoire du financement des entreprises a dû constater que les données sont partielles et qu'aucune source n'existe permettant de couvrir l'ensemble du champ de la transmission d'entreprise en France. Alors même que les entreprises doivent réaliser chaque année de nombreuses déclarations, il n'existe pas de bases de données autour de la transmission. Il n'y a même pas de définition statistique de ce concept. du dispositif Dutreil est ainsi estimé, encore en 2018, à partir de données datant de 2006 ! Le Gouvernement se heurtera aux mêmes difficultés lorsqu'il devra présenter l'étude d'impact du projet Le programme de travail de l'INSEE ne relève pas de la loi. Cependant, il m'apparaît important que les membres du Gouvernement chargés de l'économie entendent la demande du Sénat de disposer d'une meilleure connaissance statistique du tissu économique et des transmissions d'entreprise. Une

Statuant sur l'abattement de 50 %, sous conditions, sur la valeur des biens professionnels lorsque ces biens sont transmis à titre gratuit entre vifs ou par succession, le Conseil que « dans ces conditions et eu égard à l'importance de l'avantage consenti, son bénéfice est de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité entre les contribuables pour l'application du régime fiscal des droits de donation et de succession » et que, dès lors, le dispositif « ne peut être regardé dans son ensemble comme conforme à la Constitution ».

Le crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt, prévu à l'article 7, a été prorogé de deux ans, jusqu'en 2022, de manière à nous donner la possibilité d'évaluer son efficacité avant de statuer sur sa reconduction ou son abandon. Le coût de cette dépense fiscale pour les finances publiques est modéré : il n'a jamais excédé 5 millions d'euros L'assouplissement du dispositif dit « Dutreil » est conforté, d'une part, par un prolongement de droit du délai de six mois pour signer l'engagement collectif lorsque la succession n'est pas intervenue, et, d'autre part, par une prise rétroactive d'effet de l'engagement collectif à compter de la date de décès. Le principe du maintien inchangé des participations à chaque niveau d'interposition pour l'ensemble des engagements a été remplacé par celui, plus souple, du maintien du taux de participation indirecte. Le périmètre des personnes susceptibles d'exercer une fonction de direction est élargi aux cessionnaires ayant remplacé des signataires rompant leur engagement collectif en cours, en sus des nouveaux signataires ayant adhéré à un engagement collectif en cours, comme le prévoyait la proposition de loi dans

concept qui est également utilisé pour l'application de l'impôt sur la fortune immobilière et de la réduction d'impôt dite « Madelin », ainsi que pour le régime d'imposition des plus-values. Nous avons repris la définition traditionnelle tout en la complétant par la jurisprudence. C'est une première étape. Il semble néanmoins nécessaire, madame la secrétaire d'État, de reprendre les discussions avec les professionnels, abandonnées en 2014, pour préciser par circulaire les critères à mobiliser pour qualifier une animatrice. Au-delà du monde de l'entreprise, la présente proposition de loi nous invite à nous interroger sur la transmission et l'installation des agriculteurs ou des artisans. Le dispositif proposé à l'article 13 soulève de nombreuses questions quant à sa mise en oeuvre pratique. Des solutions plus satisfaisantes auraient pu être proposées par la commission des finances, mais elles seraient tombées sous le couperet de l'article 40 de la Constitution. Aucune solution plus acceptable n'ayant été trouvée au cours de la semaine écoulée, j'ai déposé un amendement de suppression de cet article, pour éviter de faire courir des risques aux potentiels bénéficiaires de cette mesure. Au moment de conclure, j'estime que le Sénat et, tout particulièrement, sa délégation aux entreprises ont fait une partie du chemin pour favoriser les transmissions d'entreprise en assouplissant les dispositifs en vigueur. Pour atteindre pleinement cet objectif, il appartient désormais à l'ensemble des acteurs qui ont vocation à conseiller et épauler les entreprises- je pense aux chambres de commerce et d'industrie, ou encore à l'agence France Entrepreneur -de faire le reste du chemin. de communiquer sur ces dispositifs qui, quand ils sont bien utilisés, permettent la continuité de l'activité économique sans nécessiter le versement de dividendes exceptionnels aux repreneurs, pour financer les charges de la donation ou de la succession.

après l'intervention de ma collègue rapporteur Christine Lavarde sur l'ensemble du texte, je me concentrerai sur le coeur de la saisine pour avis de la commission des affaires sociales, à savoir le droit à l'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise. En portant cette proposition de loi, nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart, ainsi que les membres de la délégation sénatoriale aux entreprises présidée par Élisabeth Lamure, ont souhaité apporter une réponse pragmatique à la question comment favoriser au maximum les reprises d'entreprises et, lorsque c'est possible, les reprises internes, c'est-à-dire par les salariés eux-mêmes ? Au terme de leurs auditions, ils ont conclu que le droit à l'information des salariés en cas de vente de leur entreprise, tel qu'il existe en France depuis 2014, ne fonctionne pas.

économiques, dite « loi Macron », ce dispositif demeure contre-productif, et ce pour deux raisons. En premier lieu, le délai de deux mois qu'il instaure entre la notification de l'information des salariés et la possibilité de procéder à la cession est ravageur- je pèse ce mot pour en avoir fait l'expérience ! Le caractère obligatoire et systématique de cette information peut inquiéter les salariés : lorsqu'ils reçoivent le courrier les informant de la possibilité de reprendre l'entreprise, ils ressentent généralement une profonde angoisse, et ce même lorsqu'un repreneur est pressenti. Il est ravageur aussi pour l'employeur, qui ne maîtrise pas le risque de divulgation et, à l'inverse, pâtit de la perte de confidentialité de son projet lorsqu'il a engagé des négociations avec un repreneur.

néanmoins une source de préoccupation pour les cédants potentiels, qui préfèrent bien souvent en provisionner le montant plutôt que d'informer les salariés, par crainte d'une perte de confidentialité. De l'aveu de tous les professionnels de la reprise d'entreprise- avocats, administrateurs judiciaires, experts-comptables -, ce droit à l'information n'a aucunement favorisé les reprises internes- leur nombre n'a pas progressé depuis quatre ans -, mais a entraîné de sérieuses difficultés pour certains projets de cessions

Je le dis très clairement, cette abrogation n'est pas idéologique. Je considère en effet que l'obligation d'information des salariés en cas de cession de leur entreprise peut être opportune dans certains cas, en particulier lorsqu'aucun repreneur n'est pressenti ou lorsque les salariés sont en mesure de présenter une offre de reprise concurrençant un repreneur potentiel se souciant peu de l'avenir de l'entreprise. J'ai donc proposé à la commission des affaires sociales d'émettre un avis favorable à l'amendement rétablissant l'article 15, mais à la condition que sa rédaction Si vous adoptez cet amendement modifié par le sous-amendement de notre commission, une obligation d'information sera alors instaurée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, au moment où le juge de commerce décide d'un plan de cession. À ce stade, les difficultés de l'entreprise sont connues, et il faut tout faire pour favoriser les projets de reprise. Les salariés sont alors bien placés, en raison de leur connaissance de l'entreprise, pour présenter une offre capable de convaincre le tribunal de commerce.

Mes chers collègues, nous pouvons, par cette proposition de loi, simplifier réellement la vie de nos entreprises pour favoriser leur reprise sans pour autant fragiliser les salariés. En l'état, le droit à l'information des salariés dans les PME n'est pas protecteur et ne doit pas être regardé comme un totem.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, mesdames les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi discutée Claude Nougein et Michel Vaspart, nous donne l'occasion de nous pencher sur la question de la transmission des entreprises. C'est un sujet dont la délégation aux entreprises du Sénat s'était déjà saisie il y a quelque temps, comme l'a rappelé Mme le rapporteur. Nous le savons, la transmission est un moment clef de la vie d'une entreprise, un moment charnière, souvent à haut risque. C'est également un enjeu économique important pour la pérennisation du tissu économique. Ainsi, le maintien d'un taux élevé de cession et de transmission d'entreprises est primordial, en particulier dans le contexte de vieillissement de la population des dirigeants d'entreprise en France.

faciliter les reprises d'entreprises dans notre pays, afin de soutenir l'emploi, le maintien des savoir-faire et la vitalité économique dans les territoires. C'est également un enjeu en vue de faciliter la croissance de nos PME, ce qui est l'objectif central du projet Le régime fiscal qui s'applique à la transmission, qu'elle se fasse à titre onéreux ou à titre gratuit, dans le cadre familial ou en dehors de celui-ci, ou encore dans le cas d'une transmission aux salariés, est un outil incitatif essentiel.

Les propositions d'évolution contenues dans cette proposition de loi rejoignent de façon générale les constats que nous avons établis et les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous attachons par exemple une grande importance à la transmission familiale. Comme vous le savez, le pacte Dutreil est le principal dispositif utilisé pour la transmission patrimoniale d'entreprises en France. Celle-ci est beaucoup plus faible chez nous- nous avons entendu le chiffre de 14 % -que dans les autres grands pays européens

nous proposerons l'assouplissement du dispositif Dutreil, afin de le rendre plus accessible et plus incitatif. Nous le ferons néanmoins avec le souci constant de ne pas affaiblir la robustesse juridique du dispositif. Nous avons également conscience de la nécessité de simplifier les dispositifs de soutien pour la reprise d'une entreprise par ses salariés : il s'agit d'un phénomène encore très marginal, alors qu'il fait sens dans la vie de certaines entreprises. Les dispositifs de soutien à la reprise par les salariés doivent être appréhendés dans leur globalité tant la fiscalité que la connaissance des dispositifs par les salariés. De nombreuses propositions ont été formulées en ce sens dans le cadre des travaux préparatoires du projet de loi PACTE ; nous sommes attachés à ce que tous les leviers soient mobilisés pour favoriser ce mode de transmission de façon pragmatique La modernisation de la transmission d'entreprise constitue un pan important de la réforme que nous voulons mener, mais elle n'est pas le seul enjeu qui attend nos entreprises. Avec PACTE, le Gouvernement ambitionne une réforme profonde de l'appareil productif français, de nature à soutenir la croissance et l'emploi. Nous disposons d'atouts formidables de savoir-faire et de créativité, mais ils ne sont pas suffisants dans la compétition économique mondiale nous risquons de les perdre vite si nous n'accélérons pas la transformation économique engagée. Les champs d'action sont nombreux : la création d'entreprises doit être facilitée, autant que le rebond après un échec, les freins au développement et à l'investissement doivent être levés. Il est nécessaire de mieux mobiliser l'épargne des Français, pour qu'elle bénéficie aux entreprises. Nous souhaitons également que les salariés soient mieux associés aux résultats des entreprises : c'est le sens de l'annonce par le Président de la République de la suppression du forfait social sur les accords d'intéressement dans l'ensemble des entreprises de moins de 250 salariés. La discussion d'aujourd'hui est une première occasion d'échanger sur cette problématique essentielle de la transmission. Il nous paraît néanmoins indispensable de conserver une cohérence d'ensemble

Toutefois, et bien que votre proposition de loi devance quelque peu l'appel par rapport au support législatif que nous privilégions, nous sommes ouverts à la discussion et nous remercions Mme la rapporteur des échanges que nous avons pu avoir avec elle. Vos débats contribueront certainement à enrichir les travaux préparatoires que nous menons

Or les TPE et PME emploient près de 6 millions de salariés, produisent 44 % de la valeur ajoutée du secteur marchand et composent l'essentiel du tissu économique privé.

Pourtant, au regard des enjeux d'emploi et de vitalité des territoires que la question de la transmission peut poser, il me semble que les mesures proposées se révèlent, disons, peu adéquates.

l'abrogation des obligations d'information du personnel- sujet sans rapport avec l'objectif annoncé du texte -, l'assouplissement des pactes d'actionnaire, dits « pactes Dutreil », enfin la bonification des opérations de réinvestissement des plus-values. À la lecture de ces dispositions, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, j'ai surtout envie de rappeler que, pour permettre une transmission d'entreprise qui réponde aux enjeux exposés, il est plus qu'insuffisant de proposer un catalogue d'allégements fiscaux et d'exonérations de cotisations sociales. D'autant que ces allégements semblent très ciblés. le sont même tellement que les personnes finalement concernées semblent être celles qui interviennent dans ces transmissions de la façon la plus anecdotique. Je pense notamment- mais pas seulement, j'y reviendrai -aux transmissions internes. Pour 8 % d'entre elles, il s'agit de reprises familiales. Or celles qui sont opérées par les salariés, quelle que soit la forme adoptée- société anonyme, coopérative, ou autre -représentent plus de 20 % des transmissions. Elles sont ainsi trois fois plus nombreuses que celles qui se réalisent dans le cercle familial.

part, les mettre en question, quand tant d'entreprises ne trouvent aucun repreneur ? Pourquoi, d'autre part, cette défiance à l'égard de la prise de responsabilité des salariés pour conduire l'entreprise, alors que, au contraire, il s'agit sans doute d'une des clefs du développement économique et social de notre pays ?

dont le I est par ailleurs repris et développé dans l'article 8 de la présente proposition de loi ... On ne se prend pas les pieds dans le tapis : il y a des éléments de cohérence ! Je ne doute pas que vous allez expliquer pourquoi. Ce qui manque, à mon sens, cruellement à cette proposition de loi sur la transmission d'entreprise, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ce sont des mesures à propos et à la hauteur de ses enjeux. La transmission et la pérennité de nos entreprises ne passent pas seulement, comme le préconise cette proposition de loi, par un ensemble d'arrangements fiscaux

Nous pensons qu'il existe d'autres voies. C'est pourquoi nous regrettons l'absence totale de dispositions relatives au financement bancaire dans ce texte. Lorsqu'il s'agit de financer l'activité économique, les banques ont un rôle à jouer.,

L'article 13 nous invite à favoriser les transmissions d'exploitations agricoles, commerciales ou industrielles soumises à l'imposition au taux réel. de celles qui relèvent du régime des

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, nous partageons bien entendu l'objectif de cette proposition de loi, à savoir faciliter la transmission d'entreprises, notamment dans un cadre familial. Nous le partageons, parce que nous savons que la transmission des entreprises, qui sont d'ailleurs souvent enracinées dans les territoires, est un enjeu de première importance pour soutenir l'emploi, l'activité économique et, finalement, la vitalité des territoires. Tout cela a été très bien rappelé par les auteurs de cette proposition de loi, que je tiens à remercier et dont je veux saluer l'initiative ; mon collègue Michel Canevet aura l'occasion de le développer. Je veux pour ma part ma part attirer votre attention sur le fait que, si nous partageons l'objectif de cette proposition de loi, que nous voterons, en revanche, l'outil que vous suggérez pour alléger les coûts suscite chez nous quelques inquiétudes. En effet, vous proposez d'actionner principalement le levier des niches fiscales. Une nouvelle niche est créée, une autre est prorogée, quatre sont rehaussées. Or une telle voie ne me paraît pas la mieux adaptée, et ce pour deux raisons. En premier lieu,

par méconnaissance de leur existence ou en raison de leur complexité ou de leur technicité. C'est vrai ! La Cour des comptes revient d'ailleurs régulièrement sur la question de l'efficacité des niches fiscales, qui n'est pas complètement avérée. Ainsi, alors que la complexité de notre fiscalité est régulièrement décriée, ce texte vient d'une certaine façon l'accentuer. Ce n'est pas, selon moi, un gage d'efficacité.

en commission des finances, qui a permis de sécuriser ce texte. En outre, aucune proposition n'est faite pour compenser les pertes de recettes suscitées par ces nouvelles dispositions. Or ce texte, dont six articles portent sur les niches, risque de réduire notablement nos recettes budgétaires. Je veux rappeler que, pour 2018, les niches fiscales vont coûter à l'État près de 100 milliards d'euros, soit le tiers de son budget et un montant supérieur au déficit budgétaire attendu, soit 86,7 milliards d'euros. N'oublions pas non plus que nous nous sommes engagés,

Pour le dire tel que je le pense, on ne peut pas prôner la réduction des déficits et le désendettement de la France tout en empilant des mesures dont le coût n'est pas compensé. Malgré cela, parce que ce texte envoie un signal positif en direction des TPE et PME et qu'il aborde un sujet qui mérite de trouver des réponses, nous le soutiendrons et nous le voterons. des solutions durables pour améliorer la transmission d'entreprises devront rapidement trouver leur place dans une remise à plat des aides aux entreprises, dont je rappelle qu'elles représentent aujourd'hui, toutes sphères publiques confondues, État et collectivités, quelque 140 milliards d'euros par an,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, la transmission d'entreprise constitue une réelle préoccupation et un enjeu important pour le maintien de l'emploi et de la vie dans nos territoires. Je salue donc nos collègues de la délégation aux entreprises, Claude Nougein et Michel Vaspart, pour leur travail sur ce sujet, à savoir un rapport d'information publié l'an dernier, puis la proposition de loi que nous nous avons écouté avec attention vos engagements concernant le projet de loi PACTE, mais nous discutons aujourd'hui de ce texte proposé par la délégation aux entreprises. Nous partageons le constat initial,

Or la transmission d'une entreprise est longue et complexe : elle prend en moyenne cinq ans. Il convient donc d'inciter les chefs d'entreprise à anticiper la transmission, tout en favorisant une reprise qui permette le maintien de l'activité.

Le texte que nous examinons aujourd'hui tend à harmoniser les règles fiscales indépendamment de la taille de la structure en diminuant les taux de prélèvements sur les plus-values lors des transmissions. Or, s'il nous semble tout à fait souhaitable d'exonérer un petit exploitant agricole de la Corrèze ou de la Creuse, puisse continuer à vivre lors de la transmission, il n'en va pas de même d'une grosse coopérative agro-industrielle, dont la surface financière est tout autre. Il ne s'agit que d'un exemple, mais il est bien sûr transposable à toutes les petites entreprises, partout sur le territoire. Il me semble que l'écueil à éviter, lorsque nous traitons d'un tel sujet, est de considérer une entreprise comme un simple bien, qu'on lègue ou revend. L'entreprise doit être considérée en tant qu'écosystème, avec non seulement ses infrastructures, mais également ses salariés, son impact sur le territoire et la vitalité qu'elle représente. La transmission d'une entreprise doit être entendue non comme un transfert de fonds ou une acquisition de patrimoine, mais en tant que transfert par les compétences.

Les types de transmissions que nous souhaitons favoriser sont d'une part, les transmissions familiales, lorsqu'il s'agit de continuer à faire vivre l'entreprise, et, d'autre part, la transmission aux salariés, lesquels sont, par leur position et leurs compétences, les mieux placés pour poursuivre l'activité. Le rapport d'information publié l'an dernier posait d'ailleurs cette constatation : la reprise interne constitue l'« une des reprises les plus efficaces tant en termes de pérennité de l'entreprise qu'en termes de sauvegarde des emplois À l'inverse, nous combattons un certain type de reprises par de grands groupes financiers, français ou étrangers, dont l'objectif serait de spéculer afin de réaliser une plus-value sur la liquidation de l'entreprise. Nous savons tous quel drame peuvent induire une fermeture d'entreprise et sa disparition, particulièrement dans les territoires fragilisés, où une baisse d'activité peut avoir des effets en cascade : baisse de la population, désertification des centres-villes ou centres-bourgs, baisse globale de l'activité Pour lutter contre ce genre de phénomènes, l'une des clefs est la transparence, afin de limiter les montages financiers artificiels, qui visent à acquérir une entreprise une société-écran dans le but de l'absorber. En ce sens, nous saluons la volonté de la présidente de la délégation aux entreprises, Mme Lamure, et des auteurs du texte de donner, par amendement à l'article 8, une définition claire à la notion de animatrice, ainsi que le prévoyait le texte initial. au-delà de l'insécurité juridique pour les entreprises, l'opacité qui caractérise trop souvent ce genre de sociétés. Cela permet également de distinguer une qui participe activement à l'activité de l'entreprise et peut préparer la transmission d'une d'une simple, qui aurait par exemple pour seule fin l'optimisation fiscale. Toutefois, la partie consacrée aux reprises internes, qui est affichée comme un objectif, puisque le titre IV du texte s'intitule « Favoriser les reprises internes », ne nous semble pas satisfaisante. L'une des seules avancées proposées en faveur d'une reprise par les salariés a été supprimée en commission : ainsi, l'article 15 prévoyait une obligation d'informations des salariés sur la possibilité de reprise interne au moment de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par ailleurs, l'article 14 abroge purement et simplement tout le dispositif d'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente.

nous suit, et c'est tant mieux. Nous déplorons toutefois l'absence de chiffrage des différentes mesures. Si celle-ci s'explique bien sûr en partie par le manque de données sur le sujet, il n'en demeure pas moins qu'elle fragilise le texte. Nous considérons que la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui

je tiens tout d'abord à féliciter nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart, ainsi que Mme la rapporteur, Christine Lavarde, pour leur travail au service de nos entreprises. Au fil des mois, au nom de la délégation aux entreprises, puis au sein de la commission des finances, ils ont pris la mesure d'un enjeu majeur pour notre économie, pour l'emploi local et pour le dynamisme de nos territoires. La transmission d'entreprise est en effet une composante essentielle de la vitalité d'un tissu économique. Il n'y a qu'à regarder de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, où la vigueur du « capitalisme rhénan » repose sur de grandes entreprises familiales, gérées dans une optique de long terme. On ne le dira jamais assez, le succès économique allemand repose sur le dynamisme de ses PME familiales. À titre d'exemple, 99 % des entreprises allemandes sont des PME et 95 % d'entre elles sont des entreprises familiales. Cette structure particulière du allemand permet de créer des entreprises robustes, solides, aptes à affronter la mondialisation. En Allemagne, quelque 300 000 entreprises exportent, contre trois fois moins en France. Je n'hésite pas à faire un lien entre notre déficit commercial abyssal et le poids normatif et fiscal qui pèse sur nos PME et ETI. Très bien ! Notre déficit commercial s'est creusé de près de 29 % en 2017, à plus de 62 milliards d'euros. Nous aurons beau rétablir la soutenabilité des finances publiques, si nous ne restaurons pas notre compétitivité, nous sommes condamnés au déclin économique. Face à cette urgence, madame la secrétaire d'État, nous devons enfin créer un à la française ! Nous devons soutenir les PME et ETI françaises, qui représentaient 83 % des créations d'emploi l'année dernière et qui jouent un rôle majeur d'animation de nos territoires. Nous devons en finir avec la logique des « champions nationaux », qui ne suffit pas à rendre notre économie compétitive malgré la qualité de nos fleurons industriels. Pour contribuer à la création d'un tissu robuste de PME et d'ETI, il nous faudra transformer en profondeur notre système économique dialogue social, fardeau normatif et fiscal, réforme de l'apprentissage, financement de l'économie, coopération et accompagnement à l'export ... Tous ces éléments devront être pensés dans une vision d'ensemble. Vous l'avez compris, je suis assez libéral, mais je crois que l'État stratège ne doit pas abdiquer son rôle d'animateur pour fixer les meilleures conditions de travail aux acteurs économiques. Plusieurs initiatives, parlementaire ou gouvernementale, nous sont présentées cette année dans ce sens. Cette proposition de loi en est une. Elle est le fruit d'un long travail, je l'ai dit, et elle va dans le bon sens.

Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui ? Nous connaissons très peu la réalité statistique des transmissions d'entreprises, ce qui empêche la puissance publique de mettre en place des mécanismes adaptés à la réalité. Nous sommes dans une situation où la phase de préparation des transmissions est trop peu valorisée, ce qui conduit à des démarches précipitées et parfois bâclées, au détriment de l'emploi et de l'activité. Nous sommes dans une situation où où les dispositifs fiscaux et sociaux de la transmission, dont le pacte Dutreil, ne sont plus adaptés aux réalités du terrain. À la fois trop rigides et trop peu incitatifs pour les petites entreprises, ils doivent être modernisés.

plusieurs dispositifs, notamment relatifs à la reprise interne et familiale, me semblent aller dans le sens d'une meilleure participation des salariés au destin de leur entreprise. Cette vision est conforme au voeu formulé par le général de Gaulle dans son fameux discours de Strasbourg sur la participation, où il exposait sa vision, étonnamment moderne, d'une entreprise qui trouverait son efficacité et sa justice « dans l'association, digne et féconde, et dans le partage, à visage découvert et en honnêtes actionnaires, des bénéfices et des risques Cette vision est étonnamment moderne, disais-je, car elle fait écho aux réflexions actuelles du Gouvernement sur l'objet social de l'entreprise, sans bien sûr nier que le but premier d'une entreprise est la recherche du profit, mais en prenant mieux en compte la dignité de ses salariés et la juste part d'intérêt général qui doit éclairer son action. Cette proposition de loi a une approche équilibrée de la question de la transmission d'entreprise, qui est un sujet tout à la fois économique et social. Nous souhaitons que cette approche éclaire également la construction du projet de loi PACTE. Parce que nous avons à coeur l'intérêt des chefs d'entreprise et des salariés, plus largement, parce que nous voulons transformer le tissu économique de notre pays en faveur des PME et des ETI, nous voterons en faveur de cette proposition de loi. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty. Madame la

la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise est l'aboutissement de deux ans de réflexions et d'auditions menées au sein de la délégation aux entreprises par Claude Nougein et Michel Vaspart. Il convient de les féliciter pour leur travail approfondi et méticuleux, ainsi, d'ailleurs, qu'Olivier Cadic pour son rapport d'information relatif à l'accompagnement

La transmission d'entreprise, et surtout sa réussite, est un facteur essentiel de la vitalité de notre tissu économique,

En effet, elle ne peut dépendre uniquement du flux naturel- création, disparition -, mais doit intégrer les notions de croissance, de restructuration, de fusion, d'absorption et de transmission. C'est tout un cycle de vie dont la durée est très variable, de quelques mois à plusieurs siècles. Cette difficulté d'appréhension se retrouve même en termes statistiques, comme

il est très difficile d'évaluer et de qualifier les transmissions d'entreprise. En effet, ces transmissions s'opèrent sous de multiples formes : elles peuvent être progressives ou immédiates- une reprise au tribunal, par exemple

-, d'une reprise dans le cadre d'une procédure judiciaire. Interviennent également la taille et la nature de l'activité. Je crois par conséquent que l'établissement de statistiques est appelé à se heurter à un certain nombre de difficultés,

Même si, pour les transmissions et les reprises d'entreprise, on peut relever un certain nombre de points communs dans les démarches en termes d'informations, de procédures, de règles comptables juridiques et fiscales, il n'est pas possible de modéliser la transmission d'entreprise. Le texte qui nous est proposé contient un certain nombre de dispositions qui peuvent contribuer à un taux de transmissions et à un taux de réussite de celles-ci plus élevé ; c'est d'ailleurs bien là son

avec toutes les pressions imaginables des fournisseurs, des clients, des banquiers, voire de ceux qui voulaient faire échouer cette transaction. L'entreprise est un corps vivant fragile, et la transmission est une opération délicate, dont l'issue à terme n'est pas garantie. La réussite de cette opération conditionne sa pérennité. Le texte apporte un certain nombre d'améliorations pour faciliter la transmission d'entreprise. C'est positif, mais il ne s'agit là que de mesures d'accompagnement. Au-delà de la transmission, ce texte doit s'insérer dans une démarche volontariste d'encouragement à l'entreprenariat qui se caractérise aussi par l'initiative et la prise de risques.

nous donne l'occasion de débattre aujourd'hui de la transmission des entreprises, un sujet central quand on sait que, chaque année, 60 000 entreprises sont potentiellement concernées par une cession et que, à moyen terme, 600 000 entreprises feront l'objet d'une transmission.

y est dressé et des propositions qui en émanent, les auteurs de la proposition de loi ont proposé dix-huit articles pour « simplifier, moderniser et sécuriser la transmission d'entreprises dans nos territoires

la modification de la concurrence, que certaines entreprises peinent à appréhender. En outre, en tant qu'Ultramarin,

2,6 % contre 5,5 %, soit deux fois moins. Très surprenant aussi est le calibrage juridique et financier de cette proposition de loi.

Une excellente occasion nous sera alors donnée de conduire une véritable réflexion sur le tissu économique français, sur les aides aux PME liées notamment à la question des seuils sociaux, la réforme de l'épargne retraite, la modernisation de l'épargne salariale. Madame

L'économie française a longtemps souffert d'une hypertrophie de l'État, d'un colbertisme à la française, d'une tentation protectionniste, qui a surencadré l'entreprise, ses dirigeants et ses salariés.

Le Sénat a particulièrement à coeur de jouer ce rôle de facilitateur pour créer un environnement propice au développement de l'entreprise et alléger les contraintes qui brisent tant les initiatives dans notre pays. Il faut lever les obstacles La transmission d'entreprise constitue, tout autant que la création d'entreprises, un enjeu économique majeur pour la croissance, mais aussi pour la vitalité de nos territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux.

Elles reposent le plus souvent sur des bases saines, à savoir un pragmatisme économique, une recherche de l'intérêt commun et un dialogue social sain, équilibré et permanent entre le dirigeant et les collaborateurs.

30 000 d'entre elles ne trouvent pas de repreneurs et disparaissent, bien souvent en raison d'un système fiscal lourd et complexe. On le constate sur le terrain, au contact des acteurs économiques.

Faciliter la transmission des entreprises pour assurer leur pérennité, gage du développement économique et de la création d'emploi, est un impératif pour notre pays. En ce sens, cette proposition de loi vise quatre objectifs améliorer l'accès à l'information et l'anticipation des chefs d'entreprise dans le cadre du processus de transmission ; dynamiser le financement de la transmission ; simplifier et moderniser le cadre fiscal et économique de la transmission

Le pacte Dutreil permet, sous certaines conditions, notamment un engagement de conservation, un abattement de 75 % de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, succession ou donation. il est un outil très efficace pour faciliter cette transmission, mais reste complexe dans son fonctionnement. L'assouplissement et la sécurisation du pacte Dutreil suscitent de fortes attentes. De nombreuses propositions techniques ont été formulées en ce sens ces dernières années, qu'il conviendrait de mettre enfin en oeuvre. Il s'agirait notamment de permettre la circulation des titres entre membres du pacte, sans remise en cause de l'avantage fiscal, et d'alléger les obligations déclaratives.

En contrepartie de cette exonération beaucoup plus importante, la durée totale d'engagement serait portée de quatre à cinq ans, afin de sécuriser juridiquement le dispositif et d'éviter une censure du Conseil constitutionnel. Tel est le sens de l'amendement de Mme Lamure, que j'ai cosigné. Madame la secrétaire d'État, le pacte Dutreil est un bon outil pour organiser les transmissions. Simplifions-le ! Essayons de développer son utilisation. Offrons aux entrepreneurs de notre pays une fiscalité adaptée à leurs besoins. Favorisons le maintien des entreprises dans nos territoires. Accompagnons particulièrement nos entreprises familiales, qu'il s'agisse des TPE, des PME ou des ETI.

et d'identifier leurs problèmes. Je tiens d'ailleurs à remercier nos collègues Michel Vaspart et Claude Nougein d'avoir souhaité approfondir la réflexion sur la question de la reprise et de la

mes chers collègues, c'est en juillet 2016, c'est-à-dire il y a bientôt deux ans, que le bureau de la délégation aux entreprises a décidé d'orienter les travaux de la délégation sur la reprise et la transmission d'entreprise.

et combien le coût de la transmission, même sous le régime Dutreil, mettait en péril la survie des entreprises. Nous envions la force du tissu industriel allemand, mais il faut savoir qu'il repose sur des entreprises familiales, qui ont été transmises de génération en génération et qui ont grandi au fil du temps. La France compte 83 % d'entreprises familiales, mais l'Allemagne, comme l'a rappelé Emmanuel Capus, en compte 95 % et l'Italie 93 %. Les entreprises familiales françaises n'arrivent pas à passer les générations.

Pourtant, ces entreprises ont fait la preuve de leur particulière robustesse économique. D'après une étude de PwC France, en 2016, quelque 83 % des entreprises

Ces entreprises disposent en effet de nombreux atouts : réactivité, capacité d'investissement, prise de décision à long terme. Elles sont un moteur essentiel de l'activité économique. entreprises de taille intermédiaire se distinguent en outre par leurs performances à l'export. Comme le soulignait déjà en 2010 notre collègue Bruno Retailleau, dans son rapport au Premier ministre, elles sont capables d'articuler harmonieusement le local et le global. Dès la rentrée parlementaire de septembre 2016, la délégation a donc nommé deux rapporteurs- nos collègues Michel Vaspart et Claude Nougein -pour poser un diagnostic précis sur le mal et proposer des remèdes. Après avoir entendu tous les acteurs concernés, ils ont soumis à la délégation un rapport d'information, que celle-ci a salué et adopté en février 2017. Ils concluaient à la nécessité urgente de moderniser la transmission pour sauver des emplois dans les territoires. Ce sont les préconisations de ce rapport qui sont déclinées dans la proposition de loi déposée en mars dernier. Je me félicite que ce texte soit aujourd'hui soumis au Sénat, car il vient consacrer un long travail mené au sein de notre assemblée.

La presse économique s'en est fait l'écho ces derniers jours : la transmission d'entreprise reste trop compliquée et trop risquée. Les critères du dispositif Dutreil demeurent incertains, fragilisant les pactes conclus. Les formalités à respecter sont trop contraignantes, et leur oubli peut tout invalider. Le pacte peut donc être remis en cause longtemps après la transmission, parfois douze ans après, ce qui peut avoir des conséquences financières dramatiques. Dans ce contexte, on comprend que les dirigeants hésitent à transmettre. Au-delà des questions fiscales, les dirigeants peinent à anticiper la transmission et à élaborer une vision stratégique d'avenir pour leur entreprise, afin de passer le flambeau au mieux. En interne, la reprise de l'entreprise par les salariés, qui peut être une bonne solution, n'est pas suffisamment accompagnée. C'est pour répondre à l'ensemble de ces défis que Claude Nougein et Michel Vaspart, soutenus par la majorité des membres de la délégation aux entreprises, soumettent cette proposition de loi au Sénat.

rapporteurs et d'Élisabeth Lamure, présidente de la délégation aux entreprises. Certes, nous devons encourager la création d'entreprises, mais nous devons également veiller à préserver les entreprises existantes, notamment lors de leur transmission.

S'il est difficile de voir une entreprise fermer en raison d'une trop rude concurrence, il est incompréhensible de voir une entreprise fermer faute de repreneur. Si nous nous réjouissons de la création d'associations comme « Tous repreneurs

en relevant les abattements fiscaux prévus en cas de reprise par un ou plusieurs salariés et en réduisant de quinze à cinq le nombre minimum de salariés-repreneurs requis pour bénéficier d'un crédit d'impôt.

Faciliter la vie de nos entrepreneurs afin qu'ils puissent se consacrer à leur métier peut paraître simpliste, mais c'est déjà beaucoup. Tous nous le disent, qu'ils soient commerçants, agriculteurs ou professions libérales, ils ne souhaitent pas recevoir d'aides : ils veulent pouvoir exercer leur métier. Faciliter la vie de nos entreprises, que cela plaise ou non, est une mesure sociale. L'argent public n'existant pas, nos écoles, nos hôpitaux, nos administrations dépendent de leur bonne santé. de loi, qui concerne une phase délicate de la vie des entreprises, permettra une plus grande stabilité. C'est grâce à la stabilité que de petites entreprises peuvent devenir moyennes,

n° 6. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la mesure prévue par l'article 3 porte en elle les défauts de l'ensemble de la proposition de loi. de loi. Face à un véritable problème, celui de la transmission des entreprises, résultant dans la majorité des cas du départ à la retraite du chef d'entreprise, l'article 3 prévoit une mesure d'optimisation fiscale orientée uniquement vers les cessions internes, en l'espèce les transmissions familiales. Nous savons pourtant que ce mode de transmission est le moins répandu, bien moins notamment que la reprise d'entreprises par les anciens salariés, lesquels sont les premiers concernés, dans les faits, par ce moment décisif de la vie des entreprises. Que nous propose-t-on ?

Il est trop facile d'appuyer sur le levier fiscal quand une question se pose dans le domaine économique ou social ! Quelques centaines d'euros, produits du double abattement sur la valeur d'un fonds commercial ou du matériel indispensable à l'exploitation de ce fonds, ne représentent manifestement

Ce qui compte pour la réussite d'une transmission, dont les objectifs doivent être le maintien de l'emploi et de l'activité, c'est l'implication du personnel de l'entreprise, la juste sollicitation des établissements bancaires et la définition claire des responsabilités et des rôles.

En portant de 50 % à 60 % le taux de la réduction d'impôt en cas de donation avant soixante-cinq ans, tout en ramenant de 50 % à 40 % ce taux pour les donations effectuées entre soixante-cinq et soixante-dix ans, l'article 3 de la proposition de loi vise à encourager les dirigeants d'entreprise à préparer en amont la transmission de leur société. En effet, le manque d'anticipation reste un motif d'inquiétude. Seulement 50 % des dirigeants de plus de cinquante-cinq ans ont préparé leur succession, selon l'étude BPCE de 2017. Par ailleurs, au-delà de soixante-cinq ans, les intentions de cession des dirigeants peinent à se réaliser. Au-delà de ce seuil, la dégradation du tissu productif en raison d'un sous-investissement rend la reprise particulièrement difficile. Pour répondre à M. Gabouty concernant

d'être censurée par le Conseil constitutionnel, compte tenu de l'importance de la réduction accordée, qui se cumule à une exonération d'assiette de 75 % par rapport aux règles de taxation de droit commun.

sénateur de la Corrèze, et Michel Vaspart pour leur travail très approfondi sur la transmission des entreprises. Ils connaissent très bien leur sujet, grâce à leur expérience de l'entreprise et d'élus locaux, mais également grâce à leurs travaux au sein de la délégation aux entreprises et de la commission des finances. La transmission des entreprises est un enjeu très important pour les entreprises familiales, petites, moyennes et intermédiaires, notamment dans nos territoires ruraux. Sans repreneurs d'entreprises, les territoires seraient en grande difficulté. Il faut bien sûr accompagner les entreprises, anticiper et adapter le financement de la transmission. L'article 3 prévoit de porter à 60 % le taux de réduction d'impôts lorsque le donateur est âgé de moins de

Le dispositif que nous avons proposé m'a semblé équilibré, puisque l'aménagement prévu présente l'avantage d'être incitatif, tout en étant équilibré pour les finances publiques, dans la mesure où l'augmentation du taux

Quel est l'avis de la commission ? qui a été codifié par l'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2015 et qui s'applique aux cessions réalisées depuis le 1 janvier 2016. D'après les informations de la direction de la législation fiscale, ce dispositif a été utilisé dans deux cas seulement, pour un montant d'impôt sur le revenu inférieur à 300 000 euros. L'amendement n° 21 rectifié vise à remettre en cause l'élargissement du dispositif aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 10 millions d'euros. Dans la mesure où, d'une part, le paiement échelonné de l'impôt sur les plus-values de long terme est un dispositif de bon sens, qui permet aux cédants de ne pas acquitter l'impôt avant d'avoir reçu le paiement du prix de caution, et où, d'autre part, il s'ensuit simplement un décalage de recettes pour l'État, pour un montant négligeable, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

est à M. Fabien Gay. Si plusieurs articles de faible portée ont été supprimés par la commission des finances, le présent article 8 procède à l'assouplissement du renforcement du dispositif Dutreil, dit « des pactes d'actionnaires ». Nous ne sommes pas tout à fait en présence d'une mesure gadget : ce dispositif a toujours représenté un coût significatif pour les dépenses publiques sans que son efficacité ait jamais été établie, d'autant que la participation à un pacte d'actionnaires ne présage nullement l'implication dans la gestion de l'entreprise. L'évaluation des voies et moyens chiffre le coût des opérations à 500 millions d'euros par an, au bénéfice d'un nombre de contribuables restant dans l'ordre de grandeur. La mesure a le défaut de se placer du point de vue du seul cédant et non de l'acquéreur, car la baisse des droits qui demeure dans ce texte- quelque 90 % de la valeur du fonds, selon l'article 8 -va-t-elle permettre un allégement important de la facture pour le ou les acquéreurs ? Il en va pour nous de la transmission d'entreprise comme du logement social tant que l'on ne se place pas du point de vue du cédant de l'offre, en oubliant le demandeur ou l'acquéreur, on fait fausse route. Pour la reprise d'entreprise, nous devons donc promouvoir un dispositif de crédit d'impôt pour les établissements de crédit accordant, dans la limite de 100 000 euros, des prêts sans intérêt aux repreneurs individuels ou collectifs. Pour mesurer les données du problème, on rappellera ici que l'entreprise moyenne concernée par une transmission est en général une PME de 10 à 20 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros et dont le fonds de commerce est évalué à environ 800 000 euros. Autant dire que nous attendons de notre dispositif qu'il ait un puissant effet de levier et qu'il permette effectivement le dénouement de certaines reprises, préservant ainsi l'emploi et les activités économiques. Pour son économie générale, il procède un petit peu comme le prêt à taux zéro pour les particuliers, qui a tout de même permis le développement d'une offre de logement, certes insuffisante, relativement abordable pour les primo-accédants à la propriété. Sur la foi de leur projet de reprise, de ses implications, les repreneurs pourraient donc entrer en dialogue constructif avec les établissements de crédit, fixant la quotité des prêts et les mobilisant pour le bien de l'entreprise. C'est bien ce qui nous importe. Sous le bénéfice de toutes ces observations, mes chers collègues, nous vous invitons à voter cet amendement.

suivait les auteurs de cet amendement, l'article 7 serait remplacé par une précision sur le contenu de conventions que peuvent passer les régions et les métropoles avec certains organismes financiers participant au financement de la reprise d'entreprises. Ce nouveau dispositif m'apparaît quelque peu éloigné des dispositions dont nous discutons ; par ailleurs, il ferait peser une contrainte supplémentaire sur l'action économique des collectivités locales. La commission émet donc un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

l'article 199-0 B du code général des impôts dispose que, en cas de non-respect de l'obligation de conservation des actions ouvrant droit à réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise, l'acquéreur perd seulement le bénéfice de la réduction d'impôt pour l'année de cession

code général des impôts est de garantir une stabilité d'actionnariat en contrepartie d'une réduction d'impôt. Il est considéré que la simple perte du bénéfice de la réduction d'impôt

au-delà de la durée de détention de cinq ans, les titres sont vendus à ce moment-là, on perd le bénéfice du crédit d'impôt pour la partie des emprunts qui restent à déclarer.

les PME- réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin », le PEA PME ou encore le compte PME Innovation -, qui ont tous un objectif de soutien à l'investissement dans les PME. Partant, le Gouvernement n'est favorable ni à l'article 7 ni à l'amendement n° 22

-pour les bénéficiaires qui prendraient des engagements plus stricts de conservation des titres transmis : un engagement collectif d'au moins trois ans, contre deux ans dans le dispositif actuel, et un engagement individuel d'au moins cinq ans, contre Mme la rapporteur de la commission des finances a proposé de porter à sept ans l'exigence requise pour l'engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d'exonération de 90 %. Elle estime que cet allongement de la durée requise de conservation des titres à dix ans- trois ans collectivement plus sept ans individuellement -sécuriserait la constitutionnalité du dispositif en rendant plus strictes les conditions pour en bénéficier. Elle considère en effet que le bénéfice d'un taux d'exonération fiscale à 90 combiné à la réduction d'impôt accrue pour donation avant les soixante-cinq ans du donateur risque d'être jugé excessif par le Conseil constitutionnel. Comment identifier la limite de la durée requise d'engagement total de conservation à compter de laquelle le Conseil constitutionnel avaliserait le passage d'une exonération de 75 % à 90 % des droits de mutation ? On peut observer que les auteurs de la proposition de loi, en contrepartie de l'exonération fiscale accrue, proposent déjà d'allonger notablement la durée requise de conservation des titres et, par cette augmentation, de renforcer la stabilité du capital, considération à laquelle le Conseil constitutionnel s'est déjà montré sensible. En outre, le contexte dans lequel se présente la proposition de loi- quelque 30 000 entreprises disparaissent chaque année faute d'un repreneur -fournit un motif d'intérêt général suffisant pour conférer des avantages fiscaux- préservation des emplois, pérennité de l'appareil productif. Dans sa décision de 2003, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution une exonération de 75 % assortie de six ans de stabilité du capital dans un contexte marqué par 500 000 transmissions attendues en dix ans. ans. Est-il totalement exclu qu'il donne son aval à une exonération subsidiaire- celle de 75 % demeure - de 90 %, alors que la situation est encore plus pressante qu'alors ?

En tout état de cause, le dispositif proposé par les auteurs de la proposition de loi n'octroie pas une exonération fiscale totale. Pour toutes ces raisons, le risque de censure du Conseil constitutionnel du dispositif initial proposé par les auteurs de la proposition de loi est loin d'être avéré. Cet amendement vise donc à rétablir le texte initial. Quel est l'avis de la commission ? ? Je veux revenir sur les raisons qui avaient conduit la commission des finances, lors de sa séance du 30 mai, à proposer un allongement de la durée de détention des titres relativement à l'engagement individuel. Souvent, dans cet hémicycle, le cas allemand a été cité en exemple. En effet, dans ce pays, le taux d'abattement est plus faible que le taux en vigueur chez nous, puisqu'il est de 85 % ou de 100 % selon les cas. Cependant, à la suite de la décision de la Cour de Karlsruhe, le dispositif a été durci en novembre 2016, et si le taux est bien de 85 % ou 100 %, il est accompagné d'un certain nombre de dispositifs que nous ne retrouvons pas dans le dispositif Dutreil. En effet, lorsque la valeur de l'entreprise excède 26 millions d'euros, le pourcentage d'exonération décroît progressivement pour s'éteindre au-delà de 90 millions d'euros. La transmission des biens de l'entreprise qui ne sont pas directement utiles à son activité n'est soumise à aucun régime favorable, et la condition de maintien de la masse salariale est étendue aux entreprises dont l'effectif est compris entre 6 et 20 salariés. Comme je vous l'ai dit, ces trois conditions n'ont pas d'équivalent dans le dispositif Dutreil. Par ailleurs, le taux de l'exonération partielle dont nous discutons actuellement doit être rapproché de la réduction pour âge du donateur prévue à l'article 3, que le Sénat vient de porter de 50 % à 60 %. %. Ainsi, en couplant ces deux aménagements, le taux d'imposition effectif dans le cadre d'une donation, par exemple à deux enfants, avant soixante-cinq ans d'une entreprise qui serait valorisée à 10 millions d'euros passerait de 3,1 % à 0,6 %.

du Conseil constitutionnel si la proposition de loi devait prospérer. Hier, la commission des finances a fait sien l'optimisme de la délégation aux entreprises, puisqu'elle a émis un avis favorable sur cet amendement.

même si, je le rappelle, le Gouvernement a entrepris de travailler en profondeur sur le dispositif Dutreil- il proposera des assouplissements dans le cadre du pacte -, nous ne sommes

Parce qu'elle ne pourra pas payer les droits de succession afférents à cette transmission. Au Royaume-Uni, c'est 0 % ! C'est la meilleure assurance vie que vous puissiez offrir

J'ai entendu ce qui a été dit sur une possible censure du Conseil constitutionnel. Mais là, c'est l'intérêt supérieur, c'est l'intérêt général qui est en question.

d'en faire un article à part entière du code général des impôts, en reprenant la définition qui figurait déjà dans chacun de ces trois dispositifs et en la complétant par deux dispositions nouvelles, afin de purger les principaux conflits entre l'administration fiscale et le contribuable. Il

des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature. Jusqu'à présent, la jurisprudence n'a jamais statué favorablement pour qualifier une d'animatrice sur la base

Il convient,, que soient démontrés un contrôle réel et une animation effective des filiales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, l'existence d'une convention d'animation ne saurait suffire à démontrer une influence réelle ou significative sur la conduite de la politique du groupe. De manière plus générale, compte tenu de l'importance que revêt l'appréciation des circonstances de fait dans l'appréciation du caractère animateur d'une à l'égard de son groupe, la voie législative ne nous semble pas adaptée. Selon nous, une instruction fiscale

entre société de tête, filiale immobilière chargée de la propriété des locaux commerciaux et filiales commerciales d'exploitation de chaque magasin physique, voire de magasin thématique associé- allées, jardineries, jeux, jouets, autant d'activités très importantes, qui doivent perdurer dans nos centres-villes

Certes, le Gouvernement s'est intéressé aux moyens permettant d'assouplir les conditions de remploi, dans le cadre du dispositif d'apport-cession.

Par ailleurs, ce dispositif d'expérimentation s'appliquerait également aux commerçants et aux artisans, soit à un ensemble hétérogène, rassemblant de très nombreuses petites entreprises sur lesquelles ses conséquences n'ont pas été anticipées. Le statut de l'expérimentation ne permet pas de lever ces difficultés, dans la mesure où la durée d'application du dispositif, qui inclut la période de remboursement de l'avance, soit dix ans, est inférieure à celle qui est prévue pour l'expérimentation elle-même. Il faudrait donc prévoir un mécanisme de débouclage, dans l'hypothèse où l'expérimentation ne serait pas jugée efficace.

Tout d'abord, il ne va pas de soi que la répartition de la déduction envisagée, qui réserve un tiers de la somme déduite au cédant, puisse être considérée comme concourant à l'objectif d'intérêt général. Ensuite, l'exclusion du bénéfice du dispositif des exploitations placées sous un régime fiscal autre que celui du réel agricole conduirait à traiter différemment des exploitations connaissant des situations analogues, sans justification particulière tirée de l'objectif poursuivi. Néanmoins, si ce dispositif est inopérant, il a le mérite de nous inviter à réfléchir aux moyens de fluidifier et de sécuriser les transmissions d'exploitations agricoles et artisanales. Plusieurs pistes plus simples auraient pu être explorées, comme l'allocation de moyens budgétaires supplémentaires ou l'assouplissement des critères d'attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs,

je voudrais partager avec vous un témoignage qui nous a été livré, lors de la journée de la délégation aux entreprises, par M. Olivier Meril : « Je suis dirigeant d'une entreprise de webmarketing que j'ai reprise il y a six ans. J'ai racheté mon agence en six semaines, et nous sommes passés de dix à cent dix collaborateurs. « Puis, j'ai repris une autre agence dans le même domaine. Mais, entre-temps, a été votée la loi Hamon, qui impose d'informer les collaborateurs.

au terme duquel je n'ai récupéré que trois collaborateurs sur six, soit une coquille quasiment vide. Je n'aurais pas pu reprendre la première société avec cette nouvelle loi.

de revenir à l'origine de cette proposition de loi. Le problème, si j'ai bien compris, c'est qu'un certain nombre d'activités économiques très diverses,

qui traite précisément du cas où le juge décide, à l'issue de la période d'observation, de la cession totale ou partielle de l'entreprise. D'autre part, il tend à supprimer l'obligation d'information sur l'existence de dispositifs d'aides.

de même d'ailleurs que des formations à la reprise d'entreprise. En revanche, je considère que le rôle de conseil doit être réservé aux avocats ou aux experts-comptables, lesquels pourront renvoyer vers les chambres de commerce ou les chambres de métiers, qui assistent les salariés dans leur démarche. Les aides peuvent

à la charge de l'administrateur ou du mandataire judiciaire sur la possibilité pour les salariés de soumettre une offre de reprise de l'entreprise en redressement judiciaire. Le Gouvernement considère par ailleurs qu'il n'est pas souhaitable de modifier la date à laquelle l'information est donnée. cette information soit donnée à l'ouverture de la procédure, car il importe que les salariés disposent du temps suffisant pour préparer une éventuelle offre de reprise, qui peut être déposée à tout moment au cours de la procédure. En particulier, l'obtention des financements nécessaires à la reprise peut prendre un certain temps dans le cas d'une reprise par les salariés.

de l'obligation fixée à l'article L. 1233-57-10 du code du travail d'informer les salariés, notamment sur les actions envisagées pour trouver un repreneur. proposition de loi avaient souligné que les projets de déménagement d'un établissement, y compris à quelques centaines de mètres de l'établissement initial, entraînaient des obligations liées à la recherche d'un repreneur. Il paraît donc effectivement raisonnable de les exonérer

considère que la précision proposée n'est pas souhaitable. En effet, la notion de bassin d'emploi n'a pas de définition légale et n'est pas circonscrite. Elle ne peut donc être prise comme référence dans le cadre d'une obligation légale. Cette précision est en outre inutile et source de confusion, car le code du travail précise déjà au niveau réglementaire ce que l'on entend par fermeture d'un établissement par référence à la zone d'emploi- je vous renvoie à l'article R. 1233-15 du code du travail. L'avis

vote. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe Union Centriste se réjouit également du travail réalisé par nos deux rapporteurs et de sa concrétisation dans ce texte, même si nous aurions souhaité que plus d'articles puissent être effectivement adoptés. Comme vient de l'évoquer Jean-Marc Gabouty, nous souhaitons que le projet de loi qui sera porté par le Gouvernement puisse intégrer un grand nombre des dispositions qui ont été examinées hémicycle aujourd'hui, car l'enjeu est de faciliter la reprise et la transmission d'entreprise dans notre pays. Nous avons eu des débats, notamment sur la question de l'information des salariés. J'ai pour ma part la conviction qu'un certain nombre d'opérations de reprise et de transmission doivent se faire dans la plus grande discrétion. Cela n'empêche pas, bien entendu, les salariés de s'intéresser de près à la vie de leur entreprise et de pouvoir, le cas échéant, formuler des propositions de reprise, mais ceci doit se faire dans le cadre du dialogue au sein de l'entreprise et ne nécessite pas que des

de vous remercier

à Mme le rapporteur. Pascale Gruny et moi-même souhaitons remercier la délégation aux entreprises, particulièrement Élisabeth Lamure, Michel Vaspart et Claude Nougein, d'avoir porté le sujet de la transmission des entreprises à l'ordre du jour du Sénat. Je pense que nous avons démontré aujourd'hui en débattant pendant près de quatre heures sur ce sujet que le Sénat a toujours une utilité, et peu notamment préparer les futurs projets du Gouvernement. J'ai pu constater que la rigueur, peut-être même l'orthodoxie de la commission des finances n'avaient pas su résister à l'enthousiasme des défenseurs de l'entreprise.